madame la présidente.

qui prévoit des sanctions à l'égard des salariés refusant de se soumettre aux obligations sanitaires. Ces mesures demeurent à nos yeux inadmissibles. Elles sont encore moins justifiées aujourd'hui, alors que notre pays compte 85 % de sa population majeure vaccinée. Quelle utilité présente la reconduction d'un tel système jusqu'au 28 février prochain, si ce n'est de continuer à s'inscrire dans les pas du Gouvernement en matière de police sanitaire répressive ? Tel est le sens de notre amendement.

Mme Raymonde Poncet Monge. L'article 1 D de ce texte permet à l'employeur des établissements ciblés de suspendre un salarié n'étant pas en mesure de présenter un schéma de vaccination complet.

Il paraît par conséquent excessif de prévoir la sanction d'un salarié qui démontrerait avoir accompli les premières démarches nécessaires pour se faire vacciner. Cet amendement vise donc à encadrer les dispositifs de suspension des salariés, en leur permettant de présenter

Les délits liés aux attestations frauduleuses de vaccination sont déjà passibles de lourdes sanctions, qui participent de l'instauration d'un contrôle généralisé de la population, contraire aux valeurs de notre groupe.

Cet alinéa, qui revient à remettre en question l'avis du médecin ayant fourni le certificat médical de contre-indication vaccinale, par le contrôle du médecin conseil de l'organisme d'assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée, est contraire à la déontologie de ce corps professionnel. Il suscite un sentiment de défiance injustifiée à l'égard du corps médical.

Alors même que ce test a été toléré, sous la supervision d'un professionnel de santé, durant les mois d'été, cette absence de reconnaissance soudaine de l'outil le moins onéreux pour identifier la maladie est paradoxale. S'il a été reconnu comme valable et sûr pour accéder aux établissements recevant du public (ERP), l'autotest ne saurait se voir ainsi écarté, au risque de susciter l'interrogation légitime des Français quant à l'objectif premier du Gouvernement, qui doit rester le maintien d'une situation sanitaire, et non le développement d'outils de coercition à l'encontre des Français qui ne souhaitent pas se faire vacciner.

du passe sanitaire, c'était pour assurer une disponibilité suffisante des tests, dans un contexte d'augmentation de la demande due à la généralisation du passe et compte tenu du nombre de personnes encore non vaccinées.

le dialogue préfet-maire ou même le dialogue préfet-parlementaire, ces relations ne sont pas forcément si fluides ou efficaces. Selon les territoires, ces derniers mois, la consultation des parlementaires par le préfet a pu prendre des formes plus ou moins précises et détaillées. Il apparaît plus logique que les parlementaires et les présidents des exécutifs locaux puissent émettre un avis circonstancié sur les mesures envisagées par le préfet, plutôt que d'échanger sur des pistes de manière trop générale ou, pis, sur des décisions déjà prises. Quel Défavorable.

sur le territoire de la Guyane, où la situation continue de se dégrader. Nous considérons pour notre part que, pour faire face à la dégradation de la situation, il faudrait plutôt apporter des moyens sérieux au système hospitalier de ce territoire, qui pâtissait déjà

Pour ce qui est du faible taux de vaccination relevé dans le département de la Guyane, il faudrait plutôt engager des moyens à un niveau suffisant pour mener une vaste campagne

dans les politiques publiques sanitaires. Les chiffres récents de l'assurance maladie montrent que, pour toutes les tranches d'âge, le taux de vaccination dans les communes les plus défavorisées reste significativement inférieur à celui que l'on observe dans les communes les plus favorisées

Ses conclusions doivent permettre d'accélérer la vaccination auprès des populations les plus fragiles et les plus isolées et de présenter un bilan des actions prises, afin qu'elles ne viennent pas s'ajouter à des fractures préexistantes.

par le peuple, pour le peuple, c'est bien, mais le gouvernement du rapport, par le rapport, pour le rapport, honnêtement, cela ne mène pas très loin

M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.

puisqu'il a d'ores et déjà affirmé que ni la date ni le dispositif de départementalisation ne seraient retenus avant même que l'examen du texte ne commence. De fait, ce n'est pas une surprise. Les députés ont subi le même traitement la semaine dernière, y compris ceux de votre majorité, madame la ministre.

Dans ces conditions, comment pourrait-on vous faire confiance et vous accorder encore des pouvoirs aussi importants, alors que la session parlementaire s'achève le 28 février et que vous avez déjà décidé de ne pas convoquer le Parlement dans les mois suivants ? Pourtant, il est tout à fait possible de le faire si les parlementaires vous le demandent. Nous sommes nombreux à penser que rien ne justifie aujourd'hui que l'on vous accorde ce blanc-seing. Les règles excessives meurent de leurs excès, et l'état d'urgence, comme son nom l'indique, doit répondre à une situation de crise et d'urgence, qui n'est plus Pour ma part, je refuse de banaliser un régime d'exception et je souhaiterais que l'on revienne le plus tôt possible au droit commun et aux équilibres républicains. La liberté des personnes vaccinées,

La nouvelle version du texte proposée par notre rapporteur repose sur un esprit de négociation et d'ouverture, ce qui est une voie toujours préférable aux oppositions stériles. Hélas, le Gouvernement ne semble pas disposé à entendre d'autres voix que la sienne. Pis, il nous demande de voter les yeux fermés sur un dispositif dont nous ignorons, en réalité, le contenu à venir. Certes, l'injection du vaccin n'est pas inscrite dans la loi comme étant obligatoire, mais le passe est une forme de contrainte qui a bien pour objectif de vacciner toute la population, y compris, bientôt peut-être, les enfants à partir de 5 ans.

j'estime que ce texte n'est pas légitime. J'en veux pour preuve le vote à l'Assemblée nationale, qui s'est joué à dix voix près, alors que vous détenez une confortable majorité de députés. rien ne justifie que l'on vous accorde un blanc-seing jusqu'à la fin du mois de juillet. Les Français ont respecté les règles depuis dix-huit mois : ils ont été obéissants et ont supporté les confinements, les couvre-feux, les attestations de sortie, la culpabilisation des enfants vis-à-vis de leurs grands-parents, la solitude dans les Ehpad, le télétravail et l'enseignement aux enfants par les parents, les masques, les vaccins, les passes sanitaires et toute une série d'injonctions contradictoires. Quant aux soignants, ils ont fait preuve d'un dévouement et de sacrifices qui forcent notre respect. Pour toute récompense à leur implication, on leur annonce la prolongation du passe sanitaire sans raison valable ni transparence. C'est maintenant au Gouvernement de respecter ses engagements. Je

Je comprends la préoccupation de notre collègue Leconte, parce que nous avons des compatriotes qui reçoivent des doses de vaccins dans des pays plus ou moins lointains et qui ne sont pas reconnus comme étant vaccinés quand ils arrivent en France, ces vaccins n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation scientifique et d'une autorisation de mise sur le marché dans notre pays. Toutefois, monsieur le sénateur, la mise sur le marché d'un médicament, d'un produit de santé ou d'un vaccin n'est pas une décision politique.

vise l'exclusion des personnels de crèche du champ de l'obligation vaccinale. Je le rappelle, l'obligation s'applique aux personnels exerçant dans les mêmes lieux que des professionnels de santé soumis à l'obligation.

des puériculteurs et infirmiers et du cas où ces crèches se trouvaient au sein d'un établissement de santé. Or, dans une ordonnance du 25 octobre 2021, le Conseil d'État a estimé que l'obligation vaccinale prévue par la loi du 5 août 2021 s'appliquait à l'ensemble des personnels de crèche, quand bien même celle-ci serait située hors d'un établissement de santé.

Aussi, par souci de sécurité juridique, le présent amendement vise à préciser les dispositions de l'article 12 de ladite loi, afin d'exclure expressément du champ de l'obligation vaccinale les personnels des établissements d'accueil du jeune enfant qui ne sont pas des professionnels de santé.

En cohérence, nous proposons de clarifier le régime de l'obligation vaccinale, en disposant que celle-ci ne s'applique pas aux professionnels travaillant au sein des crèches. La rédaction proposée, plus précise que les précédentes, tend à traduire autant que possible l'esprit et l'intention du législateur d'août dernier. Les deux

où les enfants en urgence vitale ne peuvent plus être soignés en raison du manque d'effectifs. On parle aujourd'hui, mes chers collègues, de tri et de perte de chance dans ces services. Je ne Si les causes de ces défections sont diverses, nombreuses et parfois anciennes, ne sous-estimons pas l'effet de la mise en oeuvre de l'obligation vaccinale des soignants. Cet amendement vise donc à abroger la suspension du contrat de travail des soignants non vaccinés, prévue par la loi du 5 août 2021. Alors que les soignants sont à bout et en nombre insuffisant, se priver d'une telle main-d'oeuvre qualifiée en pleine pandémie est une aberration. Dans mon département, des établissements de santé sont tenus de déprogrammer plus de 50 % des interventions chirurgicales, faute de personnel ; des Ehpad dépourvus d'aide-soignant gèlent des lits ; des centres médico-psychologiques renvoient leurs patients souffrant de lourds handicaps chez leurs parents, souvent âgés, qui sont dans l'impossibilité de les prendre en charge des maires déplorent la suspension de médecins généralistes, alors que les déserts médicaux sont déjà si nombreux. Les situations de ce type se comptent par milliers, laissant des malades et des familles dans une détresse extrême. Déjà, avant l'épidémie, les hôpitaux français souffraient d'un manque criant de personnel. En 2020, d'après la Fédération hospitalière de France, dans les établissements publics comme privés, il manquait 34 000 infirmières et 24 000 aides-soignants. Pis, le mercredi 13 octobre Olivier Véran estimait que l'obligation avait fonctionné, puisque seulement 15 000 soignants restaient encore non vaccinés. Qui peut se satisfaire d'un tel résultat ? Pensez-vous vraiment que l'on puisse se le permettre ? Nous devons revenir à la raison et supprimer ces sanctions, dont les conséquences sont néfastes pour les soignants et tous les usagers du service public hospitalier.

Loïc Hervé. Il s'agit d'un amendement de repli, au cas où il serait refusé de donner une valeur législative à l'instruction relative à la mise en oeuvre de l'obligation vaccinale et du passe sanitaire dans les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux de la direction générale de la cohésion sociale, en date du 20 août 2021.

d'exercer leurs fonctions en télétravail. Il est en effet surprenant de constater que des médecins ne souhaitant pas se faire vacciner et proposant d'exercer leur mission uniquement en téléconsultation se soient vu refuser cette Notre pays souffre de nombreux déserts médicaux, particulièrement en zone rurale, et nous ne pouvons pas nous permettre de perdre davantage de médecins. Dans la mesure où il n'y aura plus de contact avec les patients, l'obligation vaccinale serait injustifiée dans ce cas. Quel est l'avis de la commission de la commission des

même intention, mais leur rédaction me semble problématique en ce qu'elle lève totalement l'obligation vaccinale dans ces établissements, y compris pour les professionnels de santé, qui sont tous légalement concernés. Cela exclurait par exemple les infirmiers qui travaillent dans une crèche, ce qui n'est pas justifié.

On recense un peu moins de 8 000 suspensions prononcées pour refus vaccinal. Si celles-ci ont pu effectivement occasionner des perturbations dans certains établissements, elles ne doivent pas occulter l'esprit de responsabilité dont a fait preuve l'immense majorité, des soignants, qui se sont engagés dans une démarche vaccinale conformément à la réglementation. Les sanctions sont efficaces et proportionnées. On sait ainsi que deux tiers des professionnels suspendus ont finalement été réintégrés après s'être conformés à l'obligation vaccinale. Cela montre aussi

dans certains territoires, en particulier les Antilles et la Guyane, où la proportion de soignants vaccinés est encore de vingt points inférieure au taux national.

Il pourrait aussi entraîner des perturbations notables dans l'organisation de ces services. Le télétravail ne doit pas être utilisé pour échapper à des règles qui s'appliquent à toute la communauté de travail au sein d'une structure. Les téléconsultations ont pour objectif de faciliter l'accès aux soins de certains patients,

Le juge des référés du Conseil d'État a jugé il y a trois jours que cette lecture des dispositions de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 ne ressortait pas suffisamment de la lettre de ce texte. Le Gouvernement en a pris acte et considère que l'adoption de cet amendement apportera une réponse claire, conforme à son intention de maintenir les personnels du secteur de la petite enfance hors du périmètre de l'obligation vaccinale, dans la mesure où il ne s'agit pas de personnels soignants. En outre, le public concerné n'est pas frappé par cette pathologie.

cet article n'a pas étendu à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française les dispositions applicables au reste du territoire national. Il convient donc d'autoriser les gouvernements de ces territoires à déroger au secret médical afin de mettre en oeuvre des systèmes de traitement de données personnelles, semblables au SI-DEP TousAntiCovid. La création de systèmes de données dans le secteur de la santé relève déjà de la compétence de ces deux collectivités. Pour cette raison, l'amendement a uniquement pour objet d'encadrer la dérogation au secret médical afin de s'assurer que les systèmes mis en oeuvre localement ne dépassent pas le cadre de ce qui est strictement nécessaire à la lutte contre le covid-19.

offre moins de garanties que celle de l'amendement du Gouvernement. Après avoir initialement envisagé de recourir à une ordonnance prise sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution, le Gouvernement fait donc le choix d'inscrire cette mesure en dur dans la loi. À cet égard, je salue l'intervention

aux seules fins de lutter contre la pandémie de covid-19. Vous en avez indiqué le périmètre, madame la ministre. Néanmoins, le Gouvernement de la République a eu l'occasion de s'exprimer sur la problématique soulevée par le Pays concernant la sécurisation des dispositifs locaux de traitement d'information aux seules fins de lutter contre la covid-19. Ainsi, en séance publique à l'Assemblée nationale le 7 septembre, puis au Sénat le 9 septembre, le ministre des outre-mer s'est engagé à recourir à une à recourir à une ordonnance sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution pour créer cette base légale. Aujourd'hui, cette ordonnance n'a toujours pas été adoptée. Ce dispositif de sécurisation étant très attendu par les autorités locales, il est donc proposé au Sénat

Des données relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles pourront être partagées, le cas échéant sans le consentement des personnes intéressées. Cette faculté sera strictement limitée à la durée de l'épidémie, au plus tard jusqu'au 31 juillet 2022. Un arrêté du gouvernement de la Polynésie française, précisera, pour chaque autorité ou organisme, pour les services et les personnels concernés, les catégories de données auxquelles ils auront accès.

Gouvernement, nous contribuerons à régler un problème assez technique. La santé relève de la compétence des autorités politiques de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, tandis que le secret médical relève de la loi nationale. Pour mettre en oeuvre le système

Il s'agit de rétablir la possibilité pour les directeurs d'établissements scolaires d'accéder aux données relatives au statut vaccinal et virologique des élèves. Cet accès est indispensable pour améliorer le suivi de l'épidémie en milieu scolaire, tout en limitant autant que possible les fermetures de classes. Il est également nécessaire pour assurer un meilleur ciblage des campagnes de vaccination et de dépistage à l'école. En revanche, il ne

Celui-ci impose d'avoir connaissance des cas confirmés, d'identifier les contacts à risque et d'isoler les contacts à risque avéré. Or son application repose aujourd'hui exclusivement sur les attestations fournies par les parents d'élèves sur des circuits de communication de ces informations faisant intervenir la médecine scolaire. Ces solutions palliatives ne permettent pas de prévenir efficacement la circulation du virus dans les écoles, car les attestations parentales ne sont vérifiables qu'avec retard ou de manière aléatoire, au gré des enquêtes ponctuelles des caisses d'assurance maladie. Par ailleurs, chaque fois qu'un cas est détecté, les parents des élèves vaccinés doivent attester sur l'honneur que leur enfant n'est pas contact à risque élevé. La réitération de cette demande dès l'apparition d'un cas confirmé est incompréhensible pour les familles concernées. La connaissance du statut vaccinal ou virologique des élèves

dont le résultat est négatif de revenir en cours dès le lendemain. Pour que ce protocole puisse être mis en oeuvre, il est primordial de doter les directeurs d'établissements scolaires d'un moyen leur permettant de vérifier que seuls les élèves négatifs se présentent à l'école. J'ajoute que le droit d'accès sera mis en oeuvre dans le strict respect des règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel, en particulier des principes de minimisation et de sécurité des données. Son seul but est de contribuer le plus efficacement possible au maintien de l'ouverture des classes.

Le Gouvernement, fort des pleins pouvoirs qu'il s'arroge au fil des mois, avec un mépris total de la volonté du Sénat, présente un amendement qui, s'il était adopté, porterait une atteinte grave au secret médical à l'école primaire et secondaire.

en plus de détruire un principe fondamental de notre droit, vous négligez- une négligence de plus ! -les conséquences désastreuses à court terme : les cours d'école et les salles de classe seront plus divisées que jamais, là où elles ont besoin d'être apaisées, et vous aggraverez le retard des élèves qui rencontrent déjà des difficultés. Par ailleurs, le Syndicat national des infirmiers conseillers de santé (Snics) s'oppose au fichage des enfants et à la levée du secret médical à l'école, comme de très nombreux personnels du milieu éducatif et la grande majorité des parents, à qui vous retirez toute confiance. Vous ouvrez là une énième boîte de Pandore, aux conséquences dévastatrices. Moins d'écoles, moins de libertés, moins de protection de la vie privée : vous achevez de casser la structure qui assure encore, tant bien que mal, notre cohésion nationale. Vous confortez les bases d'une société inégalitaire, que vous avez largement contribué à développer. Apparemment, le vivre-ensemble n'est plus au programme à l'école

à plus forte raison pour les enfants ... C'est pourquoi je vous invite, mes chers collègues, à faire, à l'instar de votre serviteur, le plus mauvais accueil à cet amendement du Gouvernement.

continue de produire des effets sur les revenus des artistes et auteurs, lesquels sont perçus avec une année de décalage. Il s'agit donc de faire face aux conséquences sociales, malheureusement durables, de la crise sanitaire dans le secteur de la culture.

à Paris, lors du vote à l'urne. Les enveloppes seraient ensuite acheminées dans les chefs-lieux des circonscriptions. Quel

des agents de sécurité privés ou des fonctionnaires contrôlent l'état de santé de nos compatriotes. Je voterai contre ce texte.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous avons eu des débats respectueux, c'est la noblesse du Sénat. Comme l'a souligné Loïc Hervé, le Sénat s'apprête à adopter un texte qui a été durement amendé en commission. Je ne comprends pas que ma famille politique vienne conforter le Gouvernement dans son obstination à utiliser la situation sanitaire comme paravent à sa tentation autoritaire. Ce gouvernement nous a confinés, puis nous a vaccinés. Il a transformé les restaurateurs, les conservateurs de musée, les propriétaires de cinéma, en auxiliaires de la force publique. Il a forcé les soignants à la vaccination. Aujourd'hui, il veut nous imposer une troisième dose pour que nous conservions le passe sanitaire sans lequel nous ne pouvons plus vivre - ce même passe sanitaire dont il est démontré qu'il n'empêche pas les contaminations.

à un passe sanitaire à vie, à la vaccination obligatoire à vie. En effet, malgré toutes les atteintes à nos libertés et le nombre de personnes vaccinées, le Gouvernement agite l'épouvantail de la cinquième vague. Je ne serai pas complice de cette absurdité et, vous l'aurez compris,

présent par les Français. L'état d'urgence sanitaire, qui devait être un régime d'exception, s'insère insidieusement dans notre droit commun. La Défenseure des droits s'est d'ailleurs inquiétée de la pérennisation d'un tel régime et a mis en garde sur la difficile compréhension de certaines dispositions pouvant entraver l'exercice des droits et libertés de manière non proportionnée à l'objectif visé. Ne négligez ni les Français ni les libertés. Jusqu'à présent, nous avons été conciliants. Nous nous sommes conformés, au nom de l'intérêt général, aux directives du Gouvernement. Tant bien que mal, nous nous sommes adaptés au port du masque obligatoire, à la vaccination et aux divers confinements, reconfinements et couvre-feux. Notre résilience a des limites. Nous espérions une sortie de crise, vous nous l'aviez promis, madame la ministre, et voilà que nous nous embarquons de nouveau dans l'incertitude et la docilité. En dépit de tous les efforts fournis et des résultats obtenus face à l'épidémie, vous décidez de ne pas prendre en compte les contestations

Notre responsabilité, en tant qu'élus de la République, est de porter la voix des Françaises et des Français, lassés de l'addiction du Gouvernement aux mesures restrictives- en fait,

et c'est le troisième élément qui constitue notre identité institutionnelle, nous sommes extrêmement soucieux de proportionner les mesures de contrainte à la situation réelle

à ceux qui contestent votre dérive autoritaire et, peut-être aussi, affaiblir le consentement des Français à ces contraintes. La parole

de l'innovation qui sont tout à l'honneur d'une commission restreinte dont nous ignorions complètement qu'elle fût possible,

les libertés publiques soient préservées autant que possible, pour que les moyens du Gouvernement soient encadrés, pour que le rôle du Parlement soit respecté et que, néanmoins,

au Gouvernement les pleins pouvoirs jusqu'au mois de juillet prochain. Ce n'était pas acceptable, le Sénat ne l'a pas accepté, c'est bien ! Ce texte devait également donner aux directeurs d'établissements scolaires la possibilité d'avoir accès aux données vaccinales des enfants. Ce n'était pas acceptable, le Sénat ne l'a pas accepté, c'est bien

suite de cette intervention, j'ai été inondée de courriers, d'appels, de mails, de messages innombrables, à tel point que

des médecins généralistes, des militaires, des grands-parents, des universitaires, des avocats, des coordinateurs d'essais cliniques, des présidents de syndicats professionnels, des personnels de santé, des infirmières, des kinésithérapeutes, des sages-femmes, des journalistes, des élus locaux, des salariés, des employés, des collaborateurs des sportifs, des présidents d'association, des juges, des directeurs d'hôpitaux, des malades avec contre-indications non reconnues, des éducateurs, des retraités, des chercheurs, des collectifs de parents, des collectifs de scientifiques et de nombreuses personnes guéries de la covid-19. Tous partis confondus, tous âges confondus, ils ont exprimé leur tristesse, leur souffrance,

à prolonger les situations d'urgence, qu'elles soient, hier, terroristes ou, aujourd'hui, sanitaires. Ce n'est pas le coup d'État permanent, c'est l'état d'urgence permanent qui nous est servi aujourd'hui. Décidément, l'exercice de la démocratie est difficile dans notre pays

Qu'importe, aujourd'hui, si le rapport bénéfice-risque décroche et devient défavorable ! L'intérêt général ne peut être invoqué indéfiniment sans s'appuyer sur des analyses complètes.

Le scrutin est ouvert.